Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons donc procéder à l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale le texte qui vous est présenté est assez peu ressemblant à celui que votre assemblée a adopté en première lecture. C'est bien dommage ! L'on peut se féliciter que des points de convergence soient apparus sur certaines dispositions essentielles, ayant trait à la stratégie de transformation du système de santé ou encore à la reconnaissance de nouveaux droits pour nos concitoyens, mais ces progrès sont indissociables d'une politique d'ensemble cohérente permettant d'inscrire ces droits nouveaux dans le cadre d'une sécurité sociale durablement équilibrée. Or le texte que vous aviez adopté mettait doublement en cause l'équilibre du projet initial. En effet, il dégradait le solde prévisionnel de plus de 700 millions d'euros et portait des options incompatibles avec les engagements que le Président de la République et la majorité de l'Assemblée nationale ont pris devant les Français. J'illustrerai mon propos en trois points. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est l'un des premiers vecteurs du plan « Ma santé 2022 ». Il ne sera pas le seul puisque, comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi Santé dans le courant du premier semestre 2022. Mais il traduit d'ores et déjà un certain nombre de dispositions qui ont vocation à figurer dans une loi financière : la diversification des modes de financement, pour prendre mieux en compte la prévention et la qualité - nous commençons par l'hôpital, mais la même logique a vocation à s'appliquer aux soins de ville l'extension du champ des expérimentations ouvertes par l'article 51 de la loi de financement pour 2018, pour susciter des innovations organisationnelles ; enfin, le renforcement des dispositifs qui incitent professionnels et établissements à améliorer la pertinence de leurs actes. Ces mesures font largement consensus entre les deux chambres ; plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été adoptées conformes, ce dont le Gouvernement se félicite. Ce projet de loi traduit notre volonté politique d'une mise en oeuvre rapide des orientations du plan « Ma santé 2022 ». L'article 29 prévoit ainsi le lancement, dès le mois de janvier prochain, de deux négociations, l'une, interprofessionnelle, relative aux communautés professionnelles territoriales de santé, l'autre, avec les médecins, portant sur la création de 4 000 postes d'assistants médicaux. sociale, avec le projet de loi Santé, nous disposerons donc des outils et des financements pour mettre en oeuvre une transformation en profondeur de l'organisation des soins de proximité dans notre pays.

sociale. Pour les familles, d'abord. Nous considérons en effet qu'une politique familiale efficace et attentive est celle qui adapte ses prestations à l'évolution des besoins et de la société. Les familles avec un enfant en situation de handicap seront davantage aidées pour faire garder leur enfant. De même, l'aide à la garde sera maintenue à taux plein lorsque l'enfant atteint ses 3 ans, et ce jusqu'à sa scolarisation, car les besoins de garde restent les mêmes tant que l'enfant n'est pas entré à l'école. Les droits des futures mères travailleuses indépendantes ou agricultrices seront alignés sur ceux des salariées, tout en restant adaptés à leur spécificité professionnelle. Le Gouvernement a soutenu à cet égard le rétablissement des dispositions conformes au rapport de la députée Marie-Pierre Rixain. sur proposition des députés, les pères d'enfants prématurés bénéficieront d'un congé indemnisé pour faciliter l'organisation de la cellule familiale dans ces circonstances très particulières. Le Parlement s'apprête également à consacrer dans ce projet de loi deux avancées sociales très importantes, particulièrement pour les personnes âgées. Dès le 1 janvier prochain, le 100 % santé commencera à devenir réalité dans la vie quotidienne de tous les À compter de cette date, les tarifs de remboursement des prothèses auditives seront revalorisés de 100 euros et le tarif des prothèses entrant dans le panier de soins sera plafonné, avec un gain moyen de 100 euros À compter du 1 avril, les tarifs de certaines prothèses dentaires seront également limités, en même temps que les soins conservateurs seront revalorisés. Cette réforme est emblématique de l'orientation que nous voulons imprimer au système de santé, avec le primat donné, toujours et partout, à la prévention et à la diminution des barrières financières pour réduire les inégalités sociales de santé. Dès l'année prochaine, l'aide à la complémentaire santé fusionnera avec la CMU complémentaire. C'est un progrès social immédiat pour 1,2 million de nos concitoyens, et un progrès potentiel pour 3 millions d'entre eux, qui pourront faire valoir leur droit à une couverture intégrale de qualité. Ces deux réformes ont été menées en concertation avec les professionnels et les assureurs complémentaires. Ce que nous avons recherché, c'est l'établissement d'un partenariat de confiance qui permette de conjuguer les efforts de tous, pour garantir aux Français une couverture de qualité et un accès effectif aux soins. Cette démarche, qui privilégie la négociation et la concertation, nous la revendiquons comme un cadre permanent de méthode, qu'il s'agisse de la santé, de la retraite ou de l'autonomie dans le grand âge. Elle est à rebours, vous en conviendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, des dispositions que vous avez introduites en première lecture et qui témoignent de divergences politiques essentielles. La majorité sénatoriale a contesté le choix que nous avons fait d'une revalorisation différenciée des prestations. Mais quelle est l'alternative que vous proposez ? Un déficit accru et une vraie remise en cause des droits de nos concitoyens.

le Gouvernement vous proposera, pour l'essentiel des dispositions de financement, le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale. La sécurité sociale est le reflet de notre société, elle accompagne son évolution. Elle doit être un cadre protecteur, équitable, stable, indépendant pour l'essentiel des statuts professionnels, au sein duquel chacun organise son parcours de vie. Nous voulons assurer son équilibre et la désendetter, pour mieux la préparer aux défis démographiques de demain. Nous voulons élargir son champ, en réinvestissant massivement des domaines du soin jusqu'à présent délaissés et en créant de nouveaux droits pour les familles. Nous voulons la rendre plus universelle et plus équitable : grâce à la fusion du RSI dans le régime général, que vous avez adoptée en 2018, les travailleurs indépendants bénéficient de droits accrus et d'une qualité de service améliorée. Ils verront, à compter de l'an prochain, leur assurance maladie gérée dans les mêmes conditions que celles qui

en première lecture, notre assemblée avait abordé ce texte de façon constructive, en adoptant notamment 49 articles sans modification, soit plus de la moitié du texte transmis par l'Assemblée nationale. Néanmoins, l'existence de quelques divergences de fond avec les députés, sur lesquelles nous reviendrons, a conduit à l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 20 novembre dernier. Vous faites état, monsieur

qui tire les conséquences de la navette sur les comptes sociaux, fait apparaître un déficit du solde consolidé des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, de 200 millions au lieu de l'excédent de 400 millions d'euros affiché lors du dépôt du texte. Autrement dit, arithmétiquement, nous ne sommes plus à l'équilibre

part, de la non-soumission à la CSG et à la CRDS des revenus du capital des personnes non inscrites à la sécurité sociale française et relevant d'une sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Il s'agit, d'autre part, de l'augmentation de la part de CSG affectée à l'UNEDIC, pour compenser la suppression des contributions chômage des salariés, du fait d'un mauvais calibrage initial lors du dépôt du texte par le Gouvernement. Cette dernière mesure illustre d'ailleurs bien la confusion croissante des ressources des administrations de sécurité sociale au sens large. La volonté de faire financer par la sécurité sociale une mesure décidée par l'État

S'agissant du sort réservé aux initiatives du Sénat, l'Assemblée nationale a repris certains des amendements que nous avions adoptés en première lecture. la suppression de l'article 7 qui concernait divers avantages sociaux comme les chèques-vacances, l'alignement sur six ans de la fiscalité sur les alcools forts dans les outre-mer, la priorité donnée aux branches et organismes les plus endettés dans les transferts de déficits cumulés de l'assurance maladie et du FSV en direction de la CADES, la Caisse d'amortissement

Sur d'autres sujets, l'Assemblée nationale n'a pas rejoint la position du Sénat, mais a fait un pas vers nos propositions. Je pense en particulier au « dispositif LODEOM », sur lequel l'Assemblée nationale a sensiblement fait évoluer sa position en maintenant les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans le régime actuel d'exonération, en adoptant des dispositions spécifiques relatives à la Guyane et en élargissant les fourchettes de rémunérations éligibles aux allégements spécifiques. En revanche, les divers élargissements sectoriels des « avantages LODEOM » votés par le Sénat n'ont pas été retenus par les députés. Concernant le dispositif dit « TO-DE » relatif aux travailleurs occasionnels du secteur agricole, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, un amendement améliorer sensiblement le mécanisme de sortie progressive issu de la première lecture. Ainsi, l'exonération totale de cotisations et contributions sociales concernera les rémunérations inférieures à 1,20 SMIC en 2019 et en 2020,

L'Assemblée nationale a ainsi rétabli le quasi-gel, à savoir une hausse de 0,3 % pendant deux ans, des prestations sociales, au détriment du pouvoir d'achat des allocataires, parmi lesquels figurent en premier lieu les retraités et les familles. Elle n'a pas non plus suivi le Sénat pour ce qui concerne les mesures d'atténuation de l'effet de seuil de la CSG pour les retraités qui passeraient du taux nul au De plus, les députés ont avalisé les conséquences financières des coupes croissantes de TVA à destination de la sécurité sociale programmées par le Gouvernement à partir de 2020. Pour mémoire, elles devraient atteindre 5 milliards d'euros par an à compter de 2022, ce qui remet en cause le désendettement de la branche maladie et du FSV. Sur la branche maladie, l'Assemblée nationale a rétabli le forfait de réorientation des urgences prévu par l'article 29 sur l'initiative de M. Véran, de même que le conditionnement des prestations de maternité à une durée minimale d'interruption d'activité de huit semaines pour les travailleuses indépendantes et les non-salariées. Nous avions proposé un dispositif plus souple, mieux adapté, pour pour ne pas dégrader les indemnités du congé maternité. Au bout du compte, les différences qui subsistent entre les deux assemblées à l'issue de cette nouvelle lecture traduisent de véritables divergences, politiques et budgétaires. Dans ces conditions, il ne semble plus possible d'adopter des amendements susceptibles d'être repris par l'Assemblée nationale en lecture définitive. La commission a donc considéré qu'il était temps de constater la fin

Mais nos débats ont aussi permis de présenter des visions très différentes de l'avenir de notre protection sociale. C'est ainsi que la démocratie se nourrit de la confrontation d'opinions distinctes et opposées. Je voudrais insister sur deux points. Tout d'abord, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, il n'y a plus d'excédent, ou plus vraiment. Le solde consolidé

Tout au long des débats, les membres du groupe socialiste et républicain se sont exprimés sur deux sujets fondamentaux. Tout d'abord, nous nous sommes résolument opposés à ce que le rapporteur général de l'Assemblée nationale a pudiquement appelé la « revalorisation différenciée » des prestations sociales. En réalité, il s'agit d'un quasi-gel des pensions de retraite et d'invalidité et des allocations familiales. Nous le disons et le redisons, une telle mesure est incompréhensible et inacceptable. En miroir de la suppression de l'impôt sur la fortune, dans le contexte de mouvements de gronde et de révolte sociale sur le thème du pouvoir d'achat, alors que les inégalités continuent de se creuser dans le monde et qu'elles ne se réduisent pas dans notre pays, cette mesure induit l'appauvrissement des personnes âgées et des familles et contient les germes d'une rupture durable de notre cohésion sociale et des menaces pour notre démocratie.

sociales. Il s'agit d'une sorte de dilution des différentes branches dans ce qui serait un grand ensemble de la protection sociale incluant les retraites complémentaires et l'assurance chômage. La règle d'or de la compensation des exonérations par le budget de l'État est mise à mal. La CSG et la TVA se substituent de manière significative aux cotisations. Les excédents futurs, hypothétiques, sont préemptés par le budget de l'État. Ainsi, la loi de financement pour 2019, qui aurait pu s'inscrire dans l'histoire comme celle du retour à l'équilibre, pourrait être celle de l'amorce d'un virage vers un modèle anglo-saxon, qui limite la protection sociale publique à un filet de sécurité pour les plus démunis. Ce débat est essentiel, il doit être mené.

À ce titre, une concertation en amont des différents groupes parlementaires ne pourrait-elle pas être utile ? Je ne suis pas la seule à m'interroger, au vu des échanges qui ont eu lieu lors de la CMP. Toutefois, pour trouver un consensus, il faut être deux ! Or la quasi-unanimité de la commission des affaires sociales regrette le manque d'écoute à l'endroit des propositions faites par le Sénat.

Concernant les minima sociaux, si nous accueillons favorablement les revalorisations de l'allocation aux adultes handicapés et du minimum vieillesse, nous ne pouvons nous en satisfaire. D'une part, elles demeurent en deçà de la hausse réelle des prix ; d'autre part, les autres minima sociaux voient leurs revalorisations plafonnées à 0,3 %, bien en deçà de l'inflation.

parcellaire, notre groupe a fait le choix d'attendre les débats qui se tiendront dans le cadre du futur projet de loi de réforme des retraites, lequel offrira à tous les parlementaires l'occasion d'un travail éclairé et approfondi.

introduit par le Sénat permettait aux médecins retraités d'obtenir, sous certaines conditions, une exonération fiscale en cas de reprise d'activité en zone sous-dense. Je crois que nous avons tous pris, dans cet hémicycle, la mesure du phénomène de désertification médicale et de son amplification à venir. J'étais particulièrement favorable à une mesure permettant de redonner du temps médical dans de nombreux territoires carencés, et regrette donc beaucoup sa suppression par l'Assemblée nationale. Je salue néanmoins le maintien de l'article 41, offrant aux médecins coordonnateurs un pouvoir de prescription médicamenteuse.

et jeunes garçons contre les papillomavirus humains dans deux régions. En effet, une bonne couverture vaccinale permettrait d'éradiquer ce virus en quelques décennies seulement. Il n'y a aucune raison valable pour que les femmes françaises soient plus exposées au risque de développer un cancer du col que leurs voisines européennes. Il ne faudra donc pas hésiter à aller plus loin en fonction du bilan de cette expérimentation et à rappeler que la balance bénéfice-risque de la vaccination est bien en faveur du bénéfice. La permanence des soins a suscité des débats nombreux et nourris. Comme d'autres collègues, j'avais déposé un amendement de suppression de l'article 29 , voté à l'unanimité par le Sénat. Sur ce sujet, les arguments ont été largement développés : payer pour ne pas soigner, reporter les actes sur une médecine de ville déjà surchargée

Toutefois, le déclenchement de ces prestations est conditionné à une durée minimale d'interruption d'activité de huit semaines, ce qui n'est pas toujours possible. Cette condition pourrait conduire les femmes qui ne peuvent pas s'arrêter aussi longtemps du fait de leur profession à y renoncer. Nous regrettons donc que les arguments de notre rapporteur Catherine Deroche n'aient pas été entendus par l'Assemblée nationale. S'agissant des grossistes-répartiteurs, nous connaissons leurs difficultés à maintenir un équilibre économique. Afin d'apporter une réponse immédiate à leurs difficultés, nous avions proposé la réduction du taux de contribution sur les génériques. Des négociations sont certes en cours, mais leur issue est incertaine et une solution d'urgence doit leur être proposée.

de faire aboutir un texte de consensus, enrichi par nos deux assemblées. Nous voterons donc contre la motion tendant à opposer la question préalable.

également les mesures favorables au fonctionnement hospitalier, relatives à son financement ou à ses objectifs : plan qualité, prévention, accès aux médicaments innovants, amélioration de certains services, dont la psychiatrie. Nous sommes favorables aux

les EHPAD, avec plus de personnels infirmiers et aides-soignants. Les principales divergences se sont cristallisées autour de la sous-revalorisation des retraites, après la réforme la CSG, en 2018, mais aussi d'autres prestations, notamment familiales. Sur cette question, le Sénat était parvenu à un texte remanié, avec une revalorisation à hauteur de l'inflation, associée à un report de l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Notre groupe a voté la revalorisation des retraites et d'autres prestations sociales, tout en proposant un dispositif intermédiaire, dans un esprit de conciliation. En effet, le recul de l'âge de départ à la retraite est une vraie question, mais ce sujet sensible nécessite une concertation en amont avec les partenaires sociaux. Aussi avons-nous proposé un dispositif alternatif de revalorisation des retraites et d'autres prestations à hauteur de 1 financé par la compensation de 1,3 milliard d'euros de diverses exonérations décidées par le Gouvernement, mais non compensées, et associé à un filet de sécurité, pour préserver les retraités les plus fragiles. Nous ne pouvons que constater l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 20 novembre dernier. Les points de divergence entre les deux chambres étaient, semble-t-il, irréconciliables, en particulier sur la question des retraites. Nous regrettons l'abandon par l'Assemblée nationale de certaines des dispositions adoptées au Sénat, notamment le maintien de l'exonération de cotisations sur les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi, qui était favorable aux agriculteurs. La suppression, même progressive, en 2020, de ce dispositif serait lourde de conséquences, notamment pour les maraîchers, les arboriculteurs et les viticulteurs, dont nous nous faisons les porte-parole. Nous sommes favorables également au rétablissement des exonérations fiscales pour favoriser l'activité des médecins retraités dans les zones sous-denses de santé, pour lutter contre la désertification médicale, mais nous sommes défavorables à l'instauration d'un forfait de réorientation des patients aux urgences, qui a été supprimé par le Sénat. Néanmoins, l'Assemblée nationale a repris quelques mesures adoptées au Sénat, notamment la suppression de l'encadrement des avantages accordés par les employeurs aux salariés, la possibilité

26 000 flacons destinés à la France seraient bloqués en Inde. Nous demandons que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé puisse réagir à cette situation d'urgence. Nous signalons aussi des risques de pénurie d'autres médicaments, comme le sel de platine. Des solutions de long terme

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je veux tout d'abord exprimer mon regret que les propositions de la commission des affaires sociales de notre assemblée aient été balayées d'un revers de manche pour la plupart d'entre elles. Pourtant, notre chambre s'est efforcée d'apporter, de façon constructive, des pistes d'amélioration de notre système de santé, tout en maintenant un équilibre budgétaire.

et aux contraintes imposées à nos établissements, qui font de la gestion de la pénurie des moyens humains et logistiques un mode opératoire. Cela reste tout à fait insuffisant, compte tenu de l'activité croissante à laquelle doivent faire face les équipes soignantes, dans des conditions de travail qui se dégradent au fil des jours. Je souhaite rappeler que nos hôpitaux publics sont à bout de souffle : malgré les efforts de rationalisation et une activité stable, l'aggravation de la situation de leurs finances persiste. Force est de constater que le déficit du budget principal des hôpitaux publics a quant à lui doublé entre 2016 et 2017, passant de 470 millions d'euros à près de 1 milliard d'euros. Outre les déficits, il faut déplorer la nouvelle baisse tarifaire de 0,8 % sur les tarifs des séjours hospitaliers en 2018, ainsi que l'économie annoncée à cinq ans de 1,2 milliard sur les dépenses de personnel. également déplorer une diminution des dépenses d'investissement, qui sont passées sous le seuil de 4 milliards d'euros en 2017. Les investissements sont pourtant indispensables à l'entretien, à la rénovation des bâtiments, au renouvellement des équipements médicaux et hôteliers ou encore à l'innovation.

à la gestion des risques et aux plaintes, vous allez leur proposer un dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité, ou IFAQ, qui prévoit notamment la mise en place d'un système de malus.

qui sont en crise. Le budget alloué à votre ministère ne répond pas à ces problèmes, non plus que l'ONDAM ou le PLFSS et surtout pas l'abandon des promesses du chef de l'État sur l'arrêt des économies réalisées sur les hôpitaux. Dès lors, une question simple se pose : quel plan d'action immédiat ? Je vous ai fait part de la situation singulière, mais non exceptionnelle du service des urgences du centre hospitalier de Perpignan, dont les médecins se disent incapables de soigner les patients qui arrivent en son sein. ils tirent simplement la sonnette d'alarme pour l'ensemble des services d'urgence de notre territoire ! Et ce n'est pas le forfait de 40 euros de réorientation des patients sur la médecine de ville qui va régler la problématique de la prise en charge des patients aux urgences. Il ouvre la voie à la rémunération de l'absence d'acte. Aussi, ce PLFSS n'apporte aucune solution capable d'améliorer les conditions d'exercice des personnels soignants, qui expriment, vous le savez bien, un sentiment de malaise, alimenté par la charge et à l'organisation du travail, la répartition du temps de travail entre les charges administratives et la fonction de soins, la nature et la répartition des tâches entre les différents professionnels de santé, l'impact de la mise en place des 35 heures, l'explosion des RTT et de l'absentéisme, l'évolution du rapport aux patients, l'ampleur des réformes et des restructurations. La frustration et l'agacement chez les soignants comme chez les patients détériorent inévitablement ce qu'ils considèrent comme le pilier de leur métier, à savoir la relation humaine. Et il me semble que ce n'est pas aux personnels soignants ni aux patients d'être des variables d'ajustement ! La rémunération des infirmiers, professionnels de santé les plus nombreux en France aujourd'hui, reste toujours aussi indigne, comme le montre le panorama 2017 de l'OCDE. situation, vous annoncez la création d'une nouvelle profession médico-administrative, celle des assistants médicaux. Cependant, de leurs missions et du calendrier d'exécution ? Ne faudrait-il pas plutôt renforcer les compétences de nos infirmiers, développer et valoriser les délégations de tâches, mieux former nos personnels et transformer la formation ? Ce sont les patients qui en pâtissent avant tout : les conditions de prises en charge sont loin d'être optimales. Les personnes âgées en souffrance et en perte d'autonomie attendent souvent des heures durant sur des brancards au service des urgences. Surtout, la baisse du nombre de lits continue. Les maladies nosocomiales représentent toujours un risque. un risque. Finalement, nous assistons progressivement à une prise en charge à deux vitesses, qui est la négation de notre système de sécurité sociale né après-guerre. Nous devons nous attacher à réformer notre système plutôt qu'à le détruire. la sortie progressive d'une vision hospitalo-centrée de notre système de soins est une issue, répondant mieux aux soins de proximité, avec l'émergence notamment de pôles d'excellence, de complémentarités, de coopérations pluriprofessionnelles et davantage d'homogénéité entre pratiques publiques et privées.

Nous l'espérons, mais je crois aussi, malheureusement, que l'ensemble des signaux d'alerte qui ont été évoqués précédemment ne seront pas levés à la seule lumière de cette nouvelle, que dis-je, de cette énième loi. Cette dernière permettra-t-elle, à elle seule, de placer le patient au coeur du système et de faire de la qualité la boussole de la réforme ? nos hôpitaux sont en apnée et votre gouvernement peine à les réanimer. Notre solidarité s'étiole là où elle devrait être à son apogée. Les professionnels, qu'ils soient administratifs, médecins ou paramédicaux, ont aujourd'hui besoin d'un signal fort de votre part. Une volonté politique est nécessaire pour réformer structurellement notre système de protection sociale et pour l'adapter aux enjeux du vieillissement et de l'innovation, en préservant son principe d'universalité. Je vous le dis aujourd'hui en tant que parlementaire qui, hier, avait des responsabilités managériales dans un établissement public et au nom de mon groupe, qui votera cette question préalable. Simone Veil le soulignait, c'est sur les drames que nous subissons que « la volonté doit refaire surface, pour un monde fraternel, un monde basé sur le respect de l'homme et sa dignité.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur

la baisse de la dépense publique, avec le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, mais également une grande ambition en matière d'accompagnement, de prévention et de simplification de notre système de santé.

de taxe sur les salaires, le CITS, en baisses de cotisations patronales sur les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC, en supprimant la totalité des cotisations patronales au niveau du SMIC à compter d'octobre 2019, alors même que, l'an dernier, dans le PLFSS pour 2018, nous avions voté la suppression des cotisations maladie et chômage, augmentant, de fait, les salaires nets ou encore en exonérant de cotisations sociales les heures supplémentaires à compter du 1 septembre 2019.

mesure de justice sociale, fruit d'un engagement présidentiel à l'égard des plus précaires et des retraités. C'est un PLFSS de simplification des normes de santé, avec l'amorce d'une véritable politique du médicament, avec une profonde modification non seulement du financement des molécules innovantes, mais aussi des règles liées à l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, ou à l'autorisation temporaire d'utilisation, l'ATU. C'est enfin un PLFSS de prévention. La maladie de bon pronostic est celle que l'on n'aura pas. À ce sujet, je sais que la ministre des solidarités et de la santé, Mme Agnès Buzyn, a à coeur de faire de notre politique en matière de prévention un point fort de la politique de santé de notre pays. À ce titre, vous avez souhaité intégrer à ce PLFSS un renforcement de la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, des actions de prévention à destination des enfants et des jeunes ou encore la traduction de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement. C'est enfin un PLFSS d'avenir, qui amorce la grande réforme de notre système de santé. Je salue, ainsi, la fin, dans les hôpitaux, du « tout-tarification à l'activité », la T2A, avec la création d'un forfait pour les maladies chroniques. Nous resterons attentifs à la mise en place du dispositif, de son extension future et, surtout, de l'articulation qu'il faudra trouver entre médecine de ville et hôpital. nous est soumis est donc sérieux et novateur. Néanmoins, car il y a toujours un néanmoins, je regrette le blocage politique qui se manifeste aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle lecture. Peut-être la marche était-elle trop haute, ou les attentes trop fortes. Toutefois, je tiens à préciser que le dialogue a eu lieu. Certes, je l'avoue, je suis un peu déçu que certaines propositions du Sénat, votées souvent à l'unanimité, n'aient pas été entendues par nos collègues députés.

La ministre Annick Girardin a présenté à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, une solution pérenne pour que ces territoires, notamment la Guyane, soient également gagnants en matière de baisse de charges. Je me félicite d'ailleurs, à ce titre, que le Gouvernement consente à mettre en place un dispositif expérimental de vaccination des personnels soignants contre la grippe, conformément à l'une de nos propositions, votée ici en première lecture, qui, grâce à la navette parlementaire, va devenir un vrai dispositif, qui pourra porter ses fruits. Je suis également ravi que nous ayons supprimé l'article 7 sur la fiscalité des avantages des comités d'entreprise et qu'un travail de fond s'annonce avec les acteurs du secteur pour parvenir à sécuriser ce dispositif. enfin, à la question des retraites. Dès le départ, mes chers collègues, vous saviez que le dialogue sur cette question n'était pas possible, compte tenu de votre approche remettant en cause la grande réforme du système que nous souhaitons et que nous mettrons en place l'année prochaine. Vous nous parlez d'écoute, mais croyez-vous être audibles lorsque vous demandez toujours plus d'efforts aux actifs, et à eux seulement ? Par ailleurs, votre proposition de taxation des organismes de mutuelle aurait nécessité un travail beaucoup plus approfondi et des mois de concertation et de travail.

Même si, en commission, une motion tendant à opposer la question préalable a été votée, je veux croire que nous sommes capables de continuer à travailler ensemble sur ce PLFSS et qu'une nouvelle lecture au sein de notre assemblée peut participer à son amélioration. Nous voterons donc contre cette motion.

Pourtant, c'est à un véritable bouleversement de logique que l'on assiste avec ce budget de la sécurité sociale pour 2019. D'une part, son financement sera assuré à hauteur de 48 % par l'impôt, notamment la contribution sociale généralisée. D'autre part, il est mis fin au principe de compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales par l'État. Autrement dit, le Gouvernement va pouvoir utiliser les ressources de la sécurité sociale, payées par les assurés sociaux, pour renflouer les caisses de l'État. Cette nouvelle lecture conforte ces choix dévastateurs et témoigne d'un

À l'heure où la colère gronde partout dans le pays, où les salariés, les privés d'emploi, les jeunes, les retraités demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat et plus d'égalité et de justice sociale, il est choquant de voir les ministres de ce Gouvernement persister dans leurs choix. le secrétaire d'État, puisque, les députés de votre majorité, vous avez supprimé l'indexation des pensions sur l'indice des prix, votée par le Sénat. Comment accepter que vous supprimiez l'impôt sur la fortune, privant les caisses de l'État d'une somme de près de 4 milliards d'euros chaque année, et que vous fassiez les poches de la majorité des Françaises et des Français, non seulement en désindexant pensions de retraite, APL et allocations familiales, mais encore en augmentant la CSG

parce que, à refuser d'écouter celles et ceux qui manifestent- les gilets jaunes, les robes noires, les blouses blanches et tous les autres -, elle renforce, comme l'ensemble des membres du Gouvernement, la désespérance sociale. La colère des personnels, des patients, des élus doit déboucher sur une issue positive, aux antipodes de votre projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit, au contraire, de réaliser 910 millions d'euros d'économies supplémentaires sur le dos de l'hôpital public. Monsieur le secrétaire d'État, vous devez écouter les agents de l'hôpital de Douai, en grève depuis le 12 novembre dernier, les personnels et les patients du centre hospitalier de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, où ma collègue Cathy Apourceau-Poly s'est rendue, pour leur apporter tout son soutien, les agents du centre hospitalier de Niort, les 120 médecins de l'hôpital de Saint-Brieuc, qui ont démissionné de la commission médicale d'établissement, et les personnels des hôpitaux psychiatriques. Je vous le dis solennellement : il y a urgence à changer notre système de santé. Les personnels soignants et non soignants, les patients et les représentants d'usagers n'en peuvent plus. Il n'y aura pas de si vous vous contentez de modifier l'organisation du travail sans une enveloppe budgétaire à la hauteur des besoins ! Lors de l'examen du texte en première lecture, notre groupe avait déposé un amendement visant à l'instauration d'un moratoire sur la fermeture des hôpitaux et des maternités. avait permis d'engager un débat, à l'occasion duquel des collègues, de toutes sensibilités politiques, ont exprimé leurs inquiétudes concernant, notamment, les fermetures de maternités dans leurs circonscriptions. sans l'intervention du président de la commission, cet amendement aurait été adopté. Et que dire de la situation des urgences ? Permettez-moi, à cet instant, de revenir sur le rétablissement par l'Assemblée nationale de l'article 29, qui prévoit l'expérimentation d'un forfait de réorientation aux urgences. Tous les groupes politiques du Sénat, en dehors de celui de la majorité gouvernementale, ont voté, en première lecture, la suppression de cette mesure. Vos députés n'en ont pas tenu compte. C'est très grave, car la réorientation des malades ne peut pas fonctionner, compte tenu notamment de la pénurie des médecins. Les déserts médicaux s'étendent de plus en plus, dans les zones rurales

Les personnels ont besoin de reconnaissance et de dialogue dans les établissements. Les déclarations de Mme la ministre des solidarités et de la santé, qui a affirmé qu'elle ne fermerait aucun hôpital de proximité, ne sont pas de nature à les rassurer,

dans les territoires. Notre groupe a formulé des propositions de substitution en faveur d'un service public hospitalier fort. Il faut un plan d'urgence pour les hôpitaux et les EHPAD publics. La politique que vous menez n'est pas la solution. Elle aggrave les maux de notre système de santé. Avec l'argent que vous avez choisi de donner aux grandes entreprises, au travers du doublement du CICE, pour « booster » l'emploi- nous sommes loin du résultat visé ! -, vous auriez pu, par exemple, supprimer les franchises médicales et les participations forfaitaires et aller vers un remboursement des soins par l'assurance maladie, autant de mesures qui auraient facilité l'accès aux droits et aux soins des assurés sociaux ! L'orientation même du PLFSS 2019 discrédite le plan « Ma santé 2022 » du Gouvernement, les moyens n'étant pas au rendez-vous. À l'inverse de votre projet, qui est celui de l'étatisation de la sécurité sociale, avec le financement par l'impôt des prestations sociales, nous souhaitons élargir l'assiette des cotisations, notamment sur les revenus financiers et les entreprises. Durant tous nos débats, de droite se sont inscrits en faux contre cette étatisation, mais leurs actes ont démenti leurs propos, puisqu'ils ont non seulement voté toutes les exonérations de cotisations patronales, mais aussi reculé l'âge de départ à la retraite. Il ne suffit pas, chers collègues, d'avoir le bon diagnostic : il faut rompre avec les politiques menées

Nous avons modifié 30 articles, en avons supprimé 8 et ajouté 25. C'est donc avec mesure et bienveillance que le Sénat a travaillé, en gardant pour objectif de présenter un PLFSS à l'équilibre, ce qui fut le cas. Monsieur le secrétaire d'État, je tenais à rassurer votre collègue M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics : le Sénat est reconnu pour sa sagesse, et non pour son hypocrisie

Les premières déclinaisons qui se retrouvent dans le présent PLFSS vont globalement dans le bon sens. Certaines craintes subsistent toutefois concernant le reste à charge zéro. Nous serons vigilants

en précise le calendrier et définit des mesures d'adaptation pour diverses catégories d'employeurs qui bénéficiaient, jusqu'à présent, de dispositifs particuliers. Après examen attentif des effets de cet article, une solution a été trouvée pour le dispositif TO-DE, avec le maintien d'une exonération totale, même si elle n'est pas pérenne, jusqu'à 1,20 SMIC, à compter de 2019. Nous nous réjouissons de l'adoption de cette mesure, en nouvelle lecture,

J'ajoute que les dérives très inquiétantes du mouvement des « gilets jaunes », en particulier à La Réunion, témoignent d'une situation sociale infiniment préoccupante. préoccupante. Comme l'a souligné M. le rapporteur général, nous regrettons que le PLFSS ne soit désormais plus à l'équilibre, en raison, non pas de notre action, mais de l'adoption de deux amendements du Gouvernement. est troublante, lorsqu'on se rappelle que vous nous avez reproché l'adoption de mesures coûteuses ... Nous regrettons que l'Assemblée nationale n'ait pas suivi la position du Sénat, notamment quant à l'atténuation de l'effet de seuil de la CSG pour les retraités qui passeraient du taux nul au taux réduit de 3,8 %. %. Selon nous, le rétablissement du forfait de réorientation des urgences ne va pas non plus dans le bon sens. Cependant, certaines mesures proposées par le Sénat ont été conservées. Je pense en particulier à l'alignement sur six ans de la fiscalité sur les alcools forts dans les outre-mer sur celle qui est en vigueur dans l'Hexagone, ou encore à la possibilité de prescription du médecin coordonnateur des Sages, nous le sommes également lorsque nous légiférons en vertu de notre mandat et dans le respect de notre Constitution. Nous nous interrogeons : le Gouvernement souffrirait-il en découvrant que le Parlement, et singulièrement le Sénat, est réellement en mesure de proposer des solutions alternatives ?

Cette mesure, souhaitée par le Gouvernement et par l'Assemblée nationale, cible une nouvelle fois les mêmes personnes : les retraités. Les dommages collatéraux de la politique budgétaire du Gouvernement se révèlent très lourds socialement. Autant nous saluons l'effort accompli pour présenter un budget en équilibre, autant nous déplorons le levier budgétaire utilisé pour y arriver. Nous ne pouvons pas laisser le Gouvernement prendre pour cibles les retraités et les familles. C'est pourquoi nous avions rétabli l'indexation des pensions, que nous compensions, d'une part, en effectuant un prélèvement sur les OCAM et, d'autre part, en reportant l'âge de départ à la retraite. Ces deux mesures se justifient pleinement, et nous avons déjà dit pourquoi dans cet hémicycle. Monsieur le secrétaire votre collègue Mme Agnès Buzyn nous a expliqué il y a quelques jours que gouverner, c'est faire des choix. Je puis vous l'assurer : c'est ce que nous faisons aujourd'hui, tout comme dans l'exercice courant de nos mandats actuels et passés. mandats actuels et passés. Nous faisons notre travail et nous savons faire des choix. En réalité, le Gouvernement nous reproche de critiquer une mesure sans prendre en compte la globalité de sa politique.

S'il est vrai que nous vous rejoignons sur ces deux idées, plusieurs mesures de contraction budgétaire prennent vos annonces à contre-pied. Sur le terrain de l'emploi, les crédits baissent, alors que le nombre de chômeurs de longue durée a progressé de 133 % depuis 2007 et que le chômage des plus de cinquante ans augmente aussi. On n'en parle que trop peu ! Sur le terrain des solidarités, des réformes paramétriques amoindrissent les revalorisations annoncées.

J'ajoute que votre majorité à l'Assemblée nationale durcit cette ligne. En effet, c'est seule contre tous les autres groupes politiques qu'elle a rejeté, hier en commission, la proposition de loi

Pour en revenir au PLFSS, la recherche d'équilibre budgétaire, l'article 7 ou encore l'issue trouvée pour le dispositif TO-DE vont dans le bon sens. Toutefois, nous ne pouvons accepter que la seule mesure d'équilibre substantielle soit prise au détriment des familles et des retraités. Il s'agit tout de même de 3 milliards d'euros, et ce choix a des airs d'austérité segmentée ... Les principaux intéressés seront, cette année encore, mis à contribution. Ils se sont exprimés et marquent leur désapprobation. Ils seront dorénavant excédés. mixte paritaire n'a pas abouti. Aucun compromis n'a été trouvé, aucune mesure limitant les conséquences de la désindexation n'a été adoptée.

J'ai bien écouté l'orateur du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Il a déclaré en séance publique : « Nos oppositions au Sénat font reculer la France ».

balayée par l'Assemblée nationale. Le forfait de réorientation des urgences a déjà été évoqué. Le Premier ministre explique que le travail doit payer.

le rapporteur général l'a souligné il y a quelques instants : les différences qui demeurent entre les deux assemblées, à ce stade de l'examen du PLFSS, traduisent des divergences politiques de fond. Ces divergences portent principalement, d'une part, sur la vision que le Gouvernement semble avoir de la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale et, d'autre part, sur le choix délibéré et répété de la majorité de raboter le pouvoir d'achat des bénéficiaires de prestations sociales, à commencer par les retraités et les familles. propos de ce que vous appelez « la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale », les premiers messages que vous avez envoyés à travers ce texte sont particulièrement inquiétants. Je ne reviendrai pas sur les non-compensations massives de mesures nouvelles de diminution des ressources de la sécurité sociale qui figurent dans ce PLFSS, sinon pour rappeler qu'elles sont d'une ampleur inédite elles s'élèveront à 2,3 milliards d'euros en 2019, puis à 3,6 milliards d'euros en régime de croisière, dès 2020.

Vous noterez d'ailleurs que le Sénat a adopté ces mesures, ce qui témoigne de son ouverture au dialogue en la matière. Exactement ! Nous n'en sommes que mieux placés pour juger inacceptables d'autres mesures que contient ce PLFSS et que les députés viennent d'introduire ou de confirmer. Tel est le cas des coupes massives de TVA à destination de la sécurité sociale, qui interviendront dès 2020 et atteindront 5 milliards d'euros dès 2022. Il est tout à fait regrettable que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu l'amendement que le Sénat a adopté pour refuser une telle trajectoire financière. Tel est également le cas du nouveau rabotage de 200 millions d'euros de CSG, auquel vous venez de procéder à l'Assemblée nationale afin de financer auprès de l'UNEDIC des sommes manquantes du fait de la suppression des contributions salariales d'assurance chômage. l'a souligné en première lecture : ces coupes programmées de TVA ne correspondent à aucun principe figurant dans le rapport du Gouvernement, et encore moins à un quelconque principe qui aurait fait l'objet d'un dialogue avec le Parlement. Quant à l'affectation de CSG à l'UNEDIC, c'est encore pire : on aggrave la confusion entre les différents régimes au lieu d'introduire de la clarté et, au bout du compte, l'on fait financer par la sécurité sociale une mesure, à savoir la suppression des contributions chômage des salariés, qui ne la concerne en rien. En fait, le seul principe qui semble guider le Gouvernement, c'est le siphonage systématique de tout excédent

Si, même cette année, pour laquelle le Gouvernement a annoncé triomphalement le retour à l'équilibre de la sécurité sociale, l'on ne parvient pas à le respecter, qu'en sera-t-il à l'avenir, lorsque le symbole se sera estompé ? Au vu de ce que vous proposez, on ne peut qu'exprimer des doutes sur ce qu'il adviendra de la capacité réelle de la sécurité sociale à rembourser ses dettes, puis à se maintenir dans une situation d'équilibre à long terme qui lui évitera d'en creuser de nouvelles. Au sujet du nouveau rabotage, pour les deux années à venir, des prestations sociales, et en particulier des pensions de retraite, nous nous sommes déjà largement exprimés à l'occasion de la première lecture.

C'est ce que les mesures courageuses prises par les partenaires sociaux dans le cadre du régime complémentaire AGIRC-ARRCO invitent à faire dès 2019. Que vous le vouliez ou non, même dans un régime à points, le critère de l'âge de départ restera incontournable, au vu de l'évolution démographique et pour assurer un revenu décent aux retraités. Les exemples étrangers étudiés par notre commission le montrent bien ; autant ne pas le cacher aux Français et les familiariser d'ores et déjà avec cette idée. Cette mesure permettrait, à terme, d'équilibrer le système. Mais, puisque dans un premier temps, elle ne peut pas produire tous ses effets, nous avions également fait le choix, pour assurer l'équilibre des comptes dès 2019, de demander aux organismes complémentaires d'assurance maladie, les fameux OCAM, une contribution exceptionnelle pour ce seul exercice.

Au lieu de cela, vous avez fait le choix de vous attaquer, une nouvelle fois, aux retraités. En 2018, avec une inflation d'au moins 1,6 %, et même sans doute de 2 %, ces derniers auront non seulement connu une année blanche en termes de revalorisation, mais subi une amputation de 1,7 % de leur pension à cause de l'augmentation de la CSG. En 2019, avec une inflation prévue à 1,3 %, vous limiterez l'évolution de leur pension à 0,3 %, diminuant une nouvelle fois leur pouvoir d'achat de 1 %. Puis, vous recommencerez en 2020. Un tel acharnement n'est pas acceptable. Ce choix est tout à fait déséquilibré. Pis, avant la réforme systémique des retraites que vous envisagez, comment envoyer plus clairement le message que le niveau de vie des générations futures ne sera aucunement garanti au moment de leur départ à la retraite, et que le Gouvernement ne se gênera pas pour actionner le levier de la valeur du point ? Comme pour la trajectoire financière de la sécurité sociale, les choix que vous affichez aujourd'hui augurent mal de l'avenir. J'aurais pu évoquer d'autres sujets, par exemple la question des travailleurs occasionnels du secteur agricole- pour ce qui les concerne, nous prenons acte des avancées de l'Assemblée nationale tout en regrettant que les députés ne soient pas allés au bout de leur démarche pour rejoindre la position du Sénat

Il y a là des indices de dégradation de la qualité du dialogue entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Gouvernement au cours de cette législature. Cette situation me semble particulièrement préoccupante.

la commission des affaires sociales vous propose d'adopter cette motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cela étant,

étions conscients de ces désaccords, pourquoi déposer une motion tendant à opposer la question préalable ? En procédant ainsi, vous affaiblissez le rôle du Sénat pour deux raisons vous donnez le sentiment que l'Assemblée nationale à seule voix au chapitre, et vous ne permettez pas à notre assemblée de conduire à son terme un débat riche et constructif. Ainsi, vous donnez aux citoyens une image affaiblie, et de non de dialogue.

extrêmement grave. Le budget de la sécurité sociale devient une véritable variable d'ajustement du budget de l'État. C'est grave ; on entre dans une autre logique,

il faut peut-être leur dire exactement ce qui va se passer. Dans le rapport entre des cotisants et des pensionnés, il faudra bien trouver un juste milieu. Alors soit on se cache derrière son petit doigt,

autant en parler en toute vérité ! Cependant, l'affaire est délicate en ce moment. Quelles que soient les positions qui vont être prises, nos concitoyens ne peuvent plus les comprendre,

que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi. Je rappelle également que l'avis du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.